Nous poursuivons la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions.

l'article 30 prévoit de simplifier la procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire, de faciliter leur circulation sur le territoire national, d'étendre les compétences des agents de police judiciaire, de supprimer l'autorisation du procureur

regrettons encore une fois que la majorité sénatoriale ait mis de côté son souci affiché de défendre l'institution judiciaire.

rendu dans le cadre des chantiers de la justice : « les institutions nationales, en particulier les diverses Conférences, restent attachées à la formalisation d'un contrôle du parquet dès 24 heures, en particulier s'agissant de procédures à très fort enjeu répressif. Elles rappellent au surplus, comme celles des juridictions qui n'y sont pas favorables, que ce renouvellement constitue pratiquement la première occasion obligatoire d'un véritable compte rendu au parquet sur le déroulement de l'enquête Au-delà de vingt-quatre heures, la privation de liberté nécessite que l'intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en oeuvre. Rappelons que le procureur de la République est garant de la bonne tenue d'une garde à vue et que le parquet doit répondre de ses enquêtes. La suppression de cette obligation risque d'entraîner une prolongation de la garde à vue chaque fois que le service enquêteur le juge utile, sans véritable contrôle par l'autorité judiciaire. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d'une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, étant rappelé que cela n'induit pas un formalisme excessif ni des contraintes particulières. Quel

les auteurs de l'amendement ont satisfaction, puisque nous avons souhaité maintenir dans le texte de la commission cette obligation de présentation. Le dispositif de l'amendement vise cependant un sujet un peu différent,

madame la ministre, mes chers collègues, il convient de déplorer l'élargissement des modalités de l'enquête de flagrance prévu par le présent article. Cette évolution sera attentatoire aux libertés en raison des pouvoirs exorbitants de contrainte de la police en matière d'enquête de flagrance. La prolongation de huit jours supplémentaires

source de difficulté, causera l'affaiblissement des droits des justiciables. Il en sera de même pour ce qui concerne la faculté des enquêteurs de perquisitionner sans assentiment en matière d'enquête préliminaire pour les délits punis de trois ans de prison. Cela constitue un élargissement dangereux des pouvoirs de contrainte de la police,

par exemple, la possibilité donnée en matière d'enquête préliminaire de procéder à des interpellations domiciliaires, à la demande du parquet, ce qui n'était possible que dans le cadre d'un mandat de recherche. Un tel projet illustre la volonté gouvernementale de déséquilibre des pouvoirs accordés aux autorités, au détriment des droits des individus et de leur vie privée, ainsi que de celle de leurs proches, alors même qu'ils sont à ce stade de simples suspects. en l'absence d'urgence. L'extension dangereuse de mesures de contrainte de la police en phase d'enquête préliminaire est critiquable, de même que la logique sécuritaire de faire des exceptions un principe, en abaissant les libertés individuelles.

Mme Éliane Assassi. Nous pensons qu'en matière pénale ce texte marque un recul de la place du juge d'instruction et des droits de la défense. Il octroie aux policiers, sans garde-fou, des pouvoirs d'écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n'ont rien à voir avec le grand banditisme ou le terrorisme. Il fait ainsi entrer encore davantage l'état d'urgence dans l'État de droit. La justice repose sur le principe de la balance entre l'accusation et la défense. Sans équilibre, vous n'avez plus de justice. C'est la conception même de cette dernière qui est menacée, comme cela a déjà été été plusieurs fois indiqué, en particulier lors de l'examen des articles 28 et 29. L'article 32 étend le pouvoir des enquêteurs par l'intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de cinq ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée. Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d'être commis, n'ont aucune raison d'être étendus à un autre cadre juridique. Alors qu'une réflexion sur la restriction de ce régime dérogatoire de l'enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l'urgence serait nécessaire, le projet de loi prévoit au contraire l'extension et la banalisation de ce dispositif par deux moyens. Il étend, premièrement, la durée de la flagrance seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure

la formulation de la disposition et la confusion de l'étude d'impact ne permettant pas d'exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ce qui porterait dans ce cas le délai maximal à vingt-quatre jours. C'est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l'autorité judiciaire est à l'oeuvre.

les rapporteurs eux-mêmes s'étant interrogés dans leur rapport sur « la pertinence de l'extension, non négligeable, des durées prolongées de l'enquête de flagrance, dès lors qu'elle semble de moins en moins caractérisée par l'urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs

n° 32, l'allongement du délai de l'enquête de flagrance proposé pour les crimes nous avait paru acceptable en première lecture compte tenu de la brièveté du délai de droit commun de huit jours, souvent insuffisant pour mener à bien les enquêtes.

Alors qu'une telle présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour un avocat d'être présent lors de la perquisition pénale. Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.

ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, la présence de l'avocat, auxiliaire de justice, est une mesure de bon sens, contribuant à la transparence et au bon déroulement de la perquisition. Elle ne saurait de ce fait être perçue comme une obstruction à la procédure pénale et judiciaire. Permettant de prévenir toute dérive au cours des perquisitions, la présence de l'avocat nous semble pertinente. Le présent amendement va

Le II de l'article 32 vise à légaliser, dans le cadre d'une expérimentation menée jusqu'au 1 janvier 2022, l'enregistrement numérique des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits. Cette disposition, susceptible de porter une atteinte grave aux droits des individus, n'est pas acceptable. En effet, en pratique, les avocats seront alors dans l'impossibilité de contrôler en temps réel la procédure et de faire des observations qui

Concernant les règles relatives aux contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiants opérés sur les conducteurs, il envisage de confier aux agents de police judiciaire, les APJ, la possibilité de prendre seuls l'initiative d'un contrôle. vous le savez, mes chers collègues, en l'état du droit, l'initiative en la matière est prise soit à la suite d'une instruction du procureur de la République, soit sur l'initiative d'un officier de police judiciaire, Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints sur les instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. La mesure prévue dans cet article est donc loin d'être neutre. Le fait de confier l'initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d'un niveau de formation procédurale moindre et font l'objet d'un contrôle plus réduit, risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées. Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d'être cohérents avec les mesures que vous avez adoptées à l'article 30 concernant les réquisitions prises par les agents de police judiciaire. Il convient, à notre sens, d'en rester au niveau de garanties assuré par le droit en vigueur, en vertu duquel les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations, mais seul

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture et nous avions alors estimé que les ajustements qui étaient proposés par le texte concernant les prérogatives des agents de police judiciaire étaient

relatives aux décisions d'interdiction de correspondance.

Elle ne peut être mise en place que sous certaines conditions, notamment la reconnaissance des faits par la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de plaider-coupable à la française.

Comme nous l'avons expliqué en première lecture, l'article 36 étend le recours à une procédure qui est superficielle, qui entraîne un jugement dégradé, dont plus de six ans d'expérience n'ont pas démontré l'utilité et qui est de nature à créer de lourdes difficultés dans les quelques dossiers dans lesquels elle serait utilisée.

fait, cette mesure s'inscrit pleinement dans la philosophie que déploie ce projet de loi en matière de procédure pénale : aller vite, juger beaucoup et pour pas cher, peu importe le moyen ! Nous proposons par conséquent la suppression de l'article 36, les aménagements apportés par la commission des lois ne changeant rien à notre détermination.

est à Mme Esther Benbassa. Le présent article traite de l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants. Cette mesure a été présentée par le ministre de l'intérieur comme une réponse permettant de simplifier le travail des forces de l'ordre et de la justice et d'automatiser les peines en la matière. Le principe de l'individualisation de la peine est ici bafoué et la mesure octroie un pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre chargées d'appliquer la contravention. Elles pourront de ce fait sanctionner sans limites et au plus grand mépris des droits des personnes suspectées. En plus d'augmenter les inégalités des citoyens devant la loi, cette mesure est dénuée de toute réflexion sur les questions relatives à la santé publique pour ce qui a trait à la prévention et au traitement de l'addiction. Le seul effet de l'amende sera d'aggraver par une sanction pécuniaire une situation souvent déjà précaire : nous savons que les comportements de consommation sont diversifiés et divergent entre les milieux paupérisés et mondains. Ce dispositif, en plus d'accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l'usage des stupéfiants, semble inefficace compte tenu de l'impossibilité juridique d'appliquer une amende forfaitaire délictuelle pour les mineurs. Il sera donc dénué de tout effet de dissuasion de la consommation chez les populations les plus jeunes. Cette mesure, mes chers collègues, est quelque peu rétrograde. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 37. Englobant tous les stupéfiants, il paraîtra répressif pour les uns et laxiste pour les autres. Quel la commission est défavorable. Cet amendement tend à supprimer l'article 37, au motif qu'il aggraverait la répression de l'usage de stupéfiants, qui pourrait être sanctionné par une amende forfaitaire.

Le Gouvernement projette de réserver la cour d'assises en première instance aux crimes dits « les plus graves », à savoir ceux qui sont punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle. Il s'agit des meurtres et assassinats, ainsi que des crimes commis dans le cadre d'une récidive. Les crimes punis de vingt ans de réclusion ou moins, comme les viols et les vols criminels, seraient donc renvoyés non plus devant la cour d'assises, mais devant la cour criminelle départementale.

Ainsi, le but réel n'est pas la réduction des délais de jugement, mais la réduction budgétaire ! Pourtant, le dernier rapport de la Commission européenne sur l'efficacité de la justice, publié en 2016, est édifiant avec 64 euros par habitant et par an consacrés au système judiciaire, la France figure en bas du classement des pays européens. Cette situation aurait dû amener le Gouvernement à augmenter significativement le budget de la justice, afin que la France rattrape son retard en la matière et qu'elle réponde aux exigences exigences du droit européen. Enfin, de telles infractions seraient jugées sans la garantie et le regard d'un jury populaire, mais les peines encourues seraient les mêmes que celles que l'on attribue habituellement en cour d'assises. Pourtant, le jury est un échantillon parfaitement représentatif de la population d'un département département et le contexte sociologique et historique permet parfois de comprendre les raisons d'un passage à l'acte. En Martinique, la population est essentiellement créolophone et les mots employés n'ont pas toujours la même signification que celle qui est retenue dans l'Hexagone, même en français. La suppression des jurés au sein de notre territoire ne ferait donc qu'accroître le clivage culturel qui existe déjà entre les justiciables et leurs juges. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement tendant à la non-application de cette disposition à nos territoires.

relative aux crimes relevant de la Cour pénale internationale et au rôle du juge français à leur égard. Ces crimes sont les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes de guerre. Aujourd'hui, quatre verrous ne permettent pas aux juges français d'exercer les prérogatives qui sont les leurs en vertu de la Convention de Rome et le but de la proposition de loi votée de manière unanime par le Sénat était de lever trois d'entre eux. Nous

Un autre verrou est la double incrimination. C'est un problème, parce qu'il faudrait que l'incrimination soit la même en France et dans un certain nombre d'États qui n'ont pas du tout la même culture des droits de l'homme que notre pays. Je note toutefois

génocide la double incrimination tombe. En revanche, elle subsisterait pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ce que je regrette. Enfin, il reste la question de la résidence habituelle. Comme le disait Robert Badinter, les personnes qui sont coupables de ce type de crimes résident rarement dans un pavillon de banlieue de notre cher pays

dès lors que des personnes sont sur notre territoire et qu'elles sont coupables de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, il serait juste de les interpeller. En conclusion, je veux

L'objectif du Gouvernement est d'accélérer les procès d'assises et d'éviter ainsi la correctionnalisation de certains crimes. Un tel objectif peut paraître légitime, mais le moyen pour y parvenir est inadéquat. Depuis 1810- deux siècles ! -, les crimes sont jugés par des cours d'assises, où siège, à côté des magistrats professionnels, un jury composé de citoyens tirés au sort. Ce sont des représentants du peuple, des ouvriers, des agriculteurs, des chômeurs, des commerçants, des directeurs, des fonctionnaires Les cours d'assises sont des juridictions qui fonctionnent : entre 90 % et 95 % des accusés sont condamnés en premier ressort. Certes, toute institution est perfectible, mais les cours d'assises ne connaissent pas de dysfonctionnements majeurs qui devraient emporter leur disparition. La question des moyens qui leur sont octroyés se pose en revanche, à l'heure où les citoyens sont en recherche d'expression directe- nous le constatons tous les jours dans la rue ! Il est plus que jamais indispensable de continuer à associer le peuple, par l'intermédiaire des jurés, à l'acte de juger. Le peuple veut être plus proche des institutions ! Les jurés ne sont pas des juristes, ils apprécient le déroulement du procès, l'interrogatoire, les réactions des individus, cela avec une certaine sagesse. Pour ces raisons, le présent amendement prévoit la suppression de cette disposition incroyable,

a pour conséquence de supprimer le jury populaire pour les crimes passibles d'une peine d'emprisonnement de moins de vingt ans. Cette suppression des jurys populaires, représentatifs représentatifs de la population locale, est particulièrement malvenue dans les outre-mer, où les justiciables ont plus de mal à se reconnaître dans des juges potentiellement venus d'ailleurs

Aussi, cet amendement vise à maintenir dans les outre-mer la présence de jurés issus du même contexte culturel et social,

les procédures devant les cours d'assises sont extrêmement longues, alors même qu'il est souhaitable que la réponse pénale intervienne relativement rapidement, en particulier dans l'intérêt des victimes.

vue. Je me tiens à votre disposition pour lancer ce débat. En tout cas, j'y participerai volontiers et je suis prêt à vous démontrer, malgré le

sur dix départements volontaires, paraît-il, durera définitivement. Il y aura deux sortes de juridiction : des cours avec cinq magistrats et des cours d'assises avec trois magistrats et douze jurés.

il s'agit de remplacer les jurés par des professionnels, mais on n'est pas sûr que la procédure soit plus rapide. Ce faisant, on éloigne le peuple de l'acte de juger.

! Je comprends, monsieur le sénateur, mais il ne faut pas penser que les magistrats professionnels ne rendent pas la justice au nom du peuple français.

correctionnalisés parce que les victimes le demandent ou parce que cela permet d'obtenir un jugement plus rapide. Je vous prie de m'excuser, madame la présidente, mais j'ai tenu à répondre à M. le sénateur Fouché. J'en viens maintenant à l'amendement n° 73, qui vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna le bénéfice

Il vise à élargir l'application de l'interdiction du territoire, appelée communément la double peine, à tout étranger reconnu coupable d'un crime ou délit entraînant cinq ans ou plus d'emprisonnement. Cette interdiction de territoire est actuellement réservée aux crimes et délits les plus graves, à commencer par les actes terroristes. Ce nouvel article 43 entraînera, par exemple, l'application de la double peine à un individu auteur d'un vol de mobylette avec effraction, comme le rappelait Mme la garde des sceaux

ayant pour effet, selon nous, d'étendre de manière excessive et disproportionnée la peine d'interdiction du territoire français. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, madame Cukierman, cette mesure uniquement aux infractions commises en matière terroriste. Le fait de l'étendre à des peines punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement nous paraît exagéré. Cette généralisation

un certain électorat, sans prendre en considération jusqu'au bout l'intérêt et les conséquences des mesures que l'on propose. Comme cela a été expliqué en première lecture, le juge dispose déjà d'une large latitude pour décider de relever ou non la récidive légale. Sa décision a évidemment des conséquences sur l'ampleur de la condamnation éventuelle. La disposition introduite aura donc comme conséquence de forcer la main au juge, ce qui est contradictoire avec l'objectif affiché, que nous partageons toutes et tous, d'une grande écoute de la magistrature. Nous proposons par conséquent de supprimer cet article à l'efficacité incertaine et, surtout, comme je le disais d'entrée,

Finalement, on propose toujours plus de répression, toujours plus de prison, alors que nous savons tous que la lutte contre la délinquance ne rentre malheureusement pas dans cette équation,

sa peine. Le groupe Les Républicains entend revenir à la révocation automatique du sursis en vigueur avant 2014. Cette disposition avait été supprimée, parce qu'elle avait fait la preuve de son inefficacité et même et même de sa dangerosité. Elle pouvait en effet conduire à l'incarcération de personnes condamnées à de petites peines. Nous estimons que le présent article porte atteinte à l'important principe de l'individualisation des peines.

En effet, les articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale prévoient l'examen du dossier par le juge de l'application des peines selon la situation des personnes condamnées à des courtes incarcérations en vue de leur proposer une peine alternative à l'emprisonnement. Rappelons donc que l'individualisation de la peine est le principe en matière d'exécution des sentences et que l'incarcération doit être considérée comme le dernier recours. Ce principe, inscrit à l'article 132-1 du code pénal, est purement occulté par notre gouvernement. Pourtant, nous le savons, la courte incarcération a des effets délétères sur la personne condamnée. Elle peut également être la cause de suicide chez les personnes les plus vulnérables, à l'instar de ce jeune homme de 25 ans, condamné à une brève peine de prison pour délit de fraude

Adeline Hazan a rappelé à ce sujet que les politiques publiques doivent « avoir le courage d'instaurer un système de régulation carcérale, en s'interrogeant enfin sur le sens des très courtes peines » et en développant des mesures alternatives à l'incarcération. Nous ne pouvons que regretter le parti pris de l'exécutif et le recul net de tous nos principes fondateurs en matière de pénologie. Nous proposons en conséquence de supprimer l'article 45. Quel

45, telles que le Gouvernement les avait rédigées, et non pas telles que la commission des lois les a réécrites, sont utiles. du code de procédure pénale de deux ans à un an nous permettra de mieux assurer la vérité des peines prononcées et de rendre plus conforme

Les prisons françaises sont surpeuplées, particulièrement dans les outre-mer : on dénombrait 70 710 détenus, dont 5 108 dans les collectivités d'outre-mer au mois de juillet

L'une des intentions affichées dans les motifs de ce projet de loi est le désengorgement des prisons. Dans le contexte actuel, le renforcement du recours à des peines alternatives à la détention, à l'aménagement de peine, ainsi qu'à la libération conditionnelle constitue effectivement un enjeu essentiel. Or il existe une contradiction entre cette intention affichée et les effets des dispositions prévues, notamment, par l'article 45, lequel risque, au contraire, de renforcer la surpopulation carcérale. Le renforcement de l'aménagement des peines inférieures ou égales à un an de prison que prévoit le projet de loi constitue, certes, une avancée de principe, mais elle ne fait qu'entériner la pratique des tribunaux correctionnels. Il est très rare, en effet, voire exceptionnel, que des peines de prison d'un mois fassent l'objet d'un mandat de dépôt. Les peines d'emprisonnement de six mois à un an, sauf motivation spéciale, font déjà souvent l'objet d'un aménagement. En revanche,

L'office du juge de l'application des peines sera donc considérablement réduit. Ce magistrat dispose pourtant d'un pouvoir important en vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion des condamnés.

à M. Maurice Antiste. J'offrais au Gouvernement, ainsi qu'au rapporteur, l'occasion de se déculpabiliser d'avoir si souvent, ce soir, prononcé des avis négatifs, mais ils n'ont pas saisi la perche. C'est bien dommage ! Je fais tout de même une nouvelle tentative sur article. Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions instituant un mandat de dépôt différé, au profit d'un recours aux peines alternatives à l'incarcération. Le mandat de dépôt doit en effet demeurer une exception, justifiée par l'absolue nécessité que le condamné aille directement en prison. Or le risque du mandat de dépôt différé est que la décision d'incarcération devienne moins exceptionnelle pour les magistrats du tribunal correctionnel. Cette disposition banalise l'acte d'emprisonnement et restreint de fait, encore une fois, les possibilités d'aménagement de peine. de peine. Le Syndicat de la magistrature l'indique : « Le tribunal n'aura plus à assumer la violence de l'emprisonnement immédiat- l'émotion des proches, l'interpellation à la barre par les policiers -, mais l'incarcération sera inéluctable

l'automaticité de la réduction de peine est une règle bien établie et prise en compte par les magistrats. Rendre cette règle floue peut, à notre sens, perturber l'organisation actuelle de l'échelle des peines. Quel

d'avoir recours aux personnes morales habilitées.

Ces dispositions, qui visent à soumettre les personnes titulaires d'un permis de visite à toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l'établissement avant leur entrée en détention, ont été intégrées, en première lecture, à la suite de l'adoption d'un amendement du groupe Les Républicains. Limiter ainsi la capacité d'action de ces visiteurs- chacun pensera à l'association Genepi -est contraire à la recherche d'un bon climat lors de la détention et d'une future bonne réinsertion. Beaucoup de femmes et d'hommes reculent, à juste titre, devant ces pratiques peu conformes au respect de la dignité et de leur rôle, utile, pour la société. Nous proposons au Sénat de s'opposer enfin à ces dispositions.

à Mme Éliane Assassi. Cet amendement de suppression relève du même esprit que le précédent, défendu par Michelle Gréaume. La vie en prison se déroule dans des conditions particulièrement détestables. Nous sommes assez nombreux ici à user de notre droit de visite dans les établissements La multiplication des suicides, comme celui de ce jeune fraudeur du métro, il y a quelques jours, à Fleury-Mérogis, l'atteste. Vouloir encore durcir ces conditions sans élaborer d'alternatives est, selon nous, un non-sens et ne peut qu'amener, à terme, terme, une véritable explosion du système pénitentiaire français. Nous estimons suffisantes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent actuellement les fouilles en prison. Réduire les tensions, violences, actes illégaux en prison dépendra, en premier lieu, d'une baisse de la surpopulation carcérale et du développement de peines de substitution, ainsi que d'une nouvelle politique de réinsertion, exigeant, bien entendu, des moyens budgétaires accrus.

au Sénat de voter en faveur de cet amendement de suppression.

afin d'éviter toute confusion sur les opérateurs pouvant mener cette mission d'accompagnement renforcé. En inscrivant dans la loi l'existence d'un suivi de ces modalités par un établissement ou un service du secteur public ou associatif, il est créé une nouvelle mesure judiciaire pénale d'accompagnement éducatif spécifique qui fait défaut dans le texte présenté. En effet, le texte, tel qu'il est proposé aujourd'hui, ne rend pas obligatoire ce soutien renforcé à la parentalité au cours des droits de visite et d'hébergement qui doit pourtant être le corollaire obligatoire de ce nouveau droit, s'agissant des jeunes les plus en conflit avec la loi. Nous proposons donc un alinéa ainsi rédigé : « Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Je rappelle que les dispositions de l'article 52 reconnaissent aux parents d'un mineur qui fait l'objet d'une mesure de placement un droit de visite et d'hébergement, selon des modalités fixées par le juge des enfants. Mes collègues signataires de l'amendement proposent de préciser que le suivi de ces modalités est confié par le magistrat à un service ou à un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette précision a paru à la commission superfétatoire dans la mesure où ce suivi sera de fait

du 29 juillet 2011 avait instauré une contribution pour l'aide juridique forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance. Ce droit d'ester en justice, acheté sous la forme d'un timbre fiscal, concernait les justices judiciaire, civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale, voire administrative, à l'exception des situations de surendettement, de la saisine du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants. Cette contribution avait été créée pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue à laquelle avait été conduit le gouvernement de M. François Fillon. Elle avait été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu'elle constituait un véritable frein à l'accès au droit. Pour compenser la perte de recettes, une dotation budgétaire- sans doute insuffisante Le présent projet de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l'aide juridictionnelle. Son montant s'établirait entre 20 et 50 euros.

ce droit de timbre et nous vous proposons de persévérer dans cette voie

l'effort de cette nouvelle contribution sur les personnes assumant seules leurs frais de justice. Nos préoccupations se portent en particulier sur les justiciables qui seraient alors victimes de l'effet de seuil. À cette occasion, madame la ministre, vous nous aviez indiqué avoir engagé des négociations avec le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et la Bâtonnière de Paris, à la suite de la remise d'un rapport sur la question

Dans l'attente de solutions plus convenables, nous proposons donc la suppression de l'article 52 . Quel

Ce système serait exonératoire pour un certain nombre de personnes, puisque cette contribution ne serait pas acquittée pour plusieurs contentieux auxquels le présent article ajoute les procédures engagées par les salariés devant le conseil de prud'hommes.

Réintroduire le droit de timbre fait débat, il faut le reconnaître. Le droit de timbre peut en effet être une manière de responsabiliser les justiciables en les sensibilisant au coût de la justice et en évitant évitant des saisines abusives. Dans beaucoup de pays d'Europe, le paiement des frais de justice par le justiciable est une réalité, contrairement à ce qui se fait en France. L'introduction d'un droit de timbre peut également faire craindre, comme vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, de freiner l'accès à la justice.

Vous avez eu raison de rappeler, madame la sénatrice, que j'avais demandé à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale de la justice un rapport sur ces sujets. Il m'a été rendu. Dès le vote de la future loi, je prendrai, comme je m'y suis engagée, contact notamment avec le Conseil national des barreaux pour

d'une part, il est déjà possible pour les justiciables de bénéficier de consultations juridiques gratuites avant de solliciter l'aide juridictionnelle, d'autre part, une ambiguïté demeure sur la rémunération de cette consultation obligatoire : si elle était facturée, cela pourrait induire un coût élevé.

relative à l'aide juridique, qui, dans la réalité, n'a jamais été appliquée. L'article 52 prévoit que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Cette consultation serait rétribuée comme un acte d'aide juridictionnelle dès lors que le demandeur de l'aide remplirait les

quelques chiffres. Aujourd'hui, le dispositif fonctionne comme un système de guichet : 90 % des demandes formulées en première instance donnent lieu à une admission, alors même que ce taux est de 23 % devant la Cour de cassation, car l'aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs si aucun moyen de cassation ne peut être relevé. Cela montre l'efficacité du dispositif ! Ce système de contrôle du bien-fondé et de la recevabilité de la demande a également d'autres vertus. Il permettra d'orienter les demandeurs vers des procédures de conciliation

Des consultations juridiques gratuites sont évidemment d'ores et déjà délivrées dans le cadre des divers dispositifs d'accès au droit. Nous cherchons en outre à promouvoir le développement des consultations juridiques au sein des juridictions pour pour mieux conseiller les justiciables et favoriser le recours notamment aux modes alternatifs de règlement des différends. Il me semble que rendre

J'estime, là encore, qu'une telle orientation doit être étudiée dans le cadre de la réflexion plus globale à laquelle je me suis engagée, ne serait-ce que pour en maîtriser le coût. Je mets aux voix l'amendement n°

44. Cet amendement vise la suppression de l'article 53, qui, à mon sens, fragilise grandement la justice de proximité et l'égal accès au droit des justiciables. Ce texte instaure en effet un tribunal unique par département, ce qui va évidemment à l'encontre de la grande disparité de nos départements français. La création de ces tribunaux ne permet pas d'assurer la proximité du justiciable avec les lieux de justice. En fait, elle l'aggrave en raison du risque de suppression de ces chambres détachées, beaucoup plus faciles à fermer qu'une juridiction à part entière.

Nous proposons également la suppression de l'article 53. Dans sa version initiale, le Gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, de la création de chambres détachées visant à remplacer les tribunaux d'instance vidés de leur substance ; la commission est allée encore plus loin en réintroduisant les tribunaux de première instance. Aussi, alors que le Gouvernement n'excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, il s'agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département. Il me semble

L'article 53 procède à la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, créant ainsi le tribunal de première instance. Les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en oeuvre de cette disposition n'aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions. Pour un territoire rural et de montagne, cette situation pourrait porter gravement préjudice à l'accès des justiciables à la justice. En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de cent pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne et les territoires ruraux, la proximité des services publics est un facteur important, car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief. C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 53 et de maintenir l'organisation judiciaire actuelle.

non statutaire, sur le modèle du juge des tutelles et du juge aux affaires familiales. Il serait chargé d'une partie des contentieux traités dans les chambres détachées. Troisièmement, nous avons institué une garantie de localisation des emplois pour les fonctionnaires du greffe, soit au siège du tribunal de première instance, soit dans une chambre détachée, et nous avons mis en place un mécanisme d'encadrement

réduisons en aucune manière ni les implantations des juridictions ni même les compétences qu'elles exercent. Fort au contraire, nous garantissons le maintien de

! Nous offrons donc toutes ces garanties de maintien de vitalité sur le territoire. Il n'y aura dans les dispositions que nous proposons que des éléments qui permettront de renforcer le rôle des juridictions. Quant à la spécialisation

et collectivités d'outre-mer du champ d'application de l'article 53, lequel organise la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. En effet, alors que l'exposé des motifs de ce projet de loi prétend rapprocher la justice des justiciables, cet article conduira au contraire à les en éloigner. En outre-mer, la réduction croissante du service public de la justice contribuera, plus encore qu'ailleurs, à accroître le clivage culturel entre les institutions judiciaires et la population, au prix d'une incapacité toujours plus grande à assurer une régulation équitable et efficace des rapports sociaux. Le service public de la justice étant dans ces régions déjà suffisamment fragilisé, il semble nécessaire d'éviter de le fragiliser davantage par une réforme qui apparaît mal calibrée et dont l'objectif reste d'économiser des moyens humains supplémentaires pourtant indispensables. nous proposons de compléter cet article par un paragraphe précisant qu'il n'est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. Quel

pays. Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures conséquentes à la suppression des tribunaux d'instance et à l'extension des compétences des tribunaux de grande instance. Cette véritable refonte de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom devrait faire l'objet d'un large débat public et d'un projet de loi distinct de cette réforme éparse. Nous proposons donc, comme au sujet de l'article 53 que nous venons d'examiner, de supprimer cet article

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

et projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (procédure accélérée)